Monsieur le président,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

J'informe le Sénat que, d'une part, la commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats à l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi de loi en cours d'examen, et que, d'autre part, la commission des lois a procédé à la désignation des candidats aux éventuelles commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte commun sur le projet de loi et le projet de loi organique pour la régulation de la vie publique.

qu'on le veuille ou non, une forme de contournement du fait syndical et des capacités des syndicats à intervenir et à négocier. J'avais insisté sur le rôle spécifique des qui mérite de rester une instance autonome au regard de l'enjeu et de l'importance des sujets qu'elle traite. J'avais également

2. En effet, la mesure phare de cet article est le regroupement des institutions représentatives du personnel en une institution unique, exigence de longue date du MEDEF, qui concerne les droits fondamentaux des travailleurs pourtant reconnus par la Constitution et en particulier le Préambule de 1946 émanant directement du programme de la Résistance. La diversité de ces institutions, délégués du personnel, comités d'entreprise, CHSCT, constitue une force pour les salariés et leurs organisations. Et elles ont une histoire, comme l'a très bien rappelé hier soir notre collègue Roland Courteau. La mise en cause des CHSCT comme institutions indépendantes est une atteinte grave à ce qu'il reste du modèle social français. La santé au travail est un enjeu de société, un enjeu de civilisation. Alors que l'efficacité des CHSCT exigeait plus de moyens, plus de compétences pour veiller sur le bien-être des travailleurs, madame la ministre, vous endossez une responsabilité historique en provoquant une régression sans pareil en ce domaine. Un exemple : les CHSCT ont le pouvoir d'ester en justice, d'engager des expertises. En un mot, ils peuvent provoquer des sanctions pénales contre les patrons qui mettent en péril la santé de leurs employés- c'est sans doute à cela

plus de 1 200 meurent des suites d'une maladie ou d'accident professionnels. Des drames comme celui de l'amiante vont entraîner des dizaines de milliers de décès. Est-il digne de réduire dans ces conditions la protection de la santé des travailleurs au sein de l'entreprise ? Selon nous, c'est indigne et contraire au progrès humain.

Alors que la loi Rebsamen, qui a modifié profondément les règles du dialogue social en entreprise, date d'à peine deux ans et n'a fait l'objet d'aucun bilan, l'article 2 du projet de loi prévoit une complète refonte des règles de négociation dans l'entreprise. En fusionnant au sein d'une instance unique les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le projet de loi tend à réduire considérablement les prérogatives et les moyens dont disposent les représentants du personnel dans les entreprises. Il met par ailleurs en cause le rôle des syndicats en permettant à la nouvelle instance unique de disposer des attributions normalement dévolues aux délégués syndicaux. De telles dispositions tendent à affaiblir gravement les droits syndicaux et la représentation collective des intérêts des salariés et vont ainsi conduire à accroître le déséquilibre des relations sociales au sein de l'entreprise.

qu'il s'agisse de la création d'une instance unique de représentation du personnel dans l'entreprise, mais également de la revalorisation des parcours syndicaux au sein de l'entreprise et de la reconnaissance des compétences acquises dans ce cadre.

pourquoi fusionner les trois instances d'information et de consultation que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel ? Eh oui ! Et pourquoi la plupart des pays n'ont-ils pas autant d'instances pour représenter le personnel ? L'enjeu de cette

il y a un lieu, un moment et des interlocuteurs pour parler de la marche des affaires, la marche de l'entreprise, l'organisation de l'entreprise ; il y a un autre lieu, un autre temps et souvent d'autres interlocuteurs pour parler des conditions de travail, de la sécurité et de la santé au travail

Elle disposerait d'un budget de fonctionnement propre. À partir d'une certaine taille, à définir, et dans les secteurs à haut risque, il faut probablement prévoir d'emblée qu'elle ait une sous-commission qui se concentre plus sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, car il y a beaucoup de matière à discuter. Autant le faire dès maintenant ! Le fait de fusionner au-dessus va apporter beaucoup plus de prévention, car vous discuterez de l'organisation et donc de la prévention.

j'ai confié récemment à Jean-Dominique Simonpoli, directeur général de l'association Dialogues, une mission pour recenser les pratiques les plus innovantes et avancées des branches et des entreprises en matière de parcours syndicaux et nous faire des propositions opérationnelles, en liaison avec tous les partenaires sociaux, et concrètes dans ce sens. Il rendra ses conclusions dans quelques jours et ces propositions ont vocation à nourrir ce qui sera dans les ordonnances. Enfin, la discrimination syndicale existe aujourd'hui, même si nous n'avons que peu de données

de la discrimination syndicale, qui fait partie des conditions d'un dialogue serein, chacun le comprendra. Voilà quelques éléments d'éclairage issus de la concertation avec les partenaires sociaux dont je voulais vous faire part pour nourrir vos débats.

les formations proposées par les différentes organisations syndicales représentatives dans l'ensemble des entreprises tiennent compte des instances représentatives dans lesquelles siègent leurs mandants pour leur donner droit à une formation.

au-delà de mon parcours professionnel, j'ai eu à gérer 3 500 salariés, 22 centres, qui dépendaient de secteurs totalement différents, secteur privé, secteur médico-social. En travaillant

en quoi ce regroupement est une avancée. Pour moi, c'est une véritable régression

La volonté de fusionner l'ensemble va certainement poser beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, dans les entreprises, les salariés subissent les exigences de plus en plus importantes des clients,

les instances de représentation du personnel. Il n'est pas question que ces fonctions ne soient plus représentées. Il y a déjà des entreprises qui pratiquent cette représentation groupée. Je pense, par exemple, à l'entreprise Solvay,

à votre raisonnement, car il faut en parler et si on n'en parle pas maintenant vous ratifierez un dispositif auquel vous n'aurez pas participé.

qu'une seule structure qui s'intéresse à l'économie de l'entreprise, à la gouvernance, s'occupera mieux des problèmes de santé qu'une structure spécifique qui a l'habitude de traiter ces dossiers

une réalité dans tous les domaines de l'activité économique. Les contraintes économiques écrasent toutes les autres considérations. Ne pas sanctuariser les questions d'hygiène, de sécurité et de santé au travail, c'est risquer de les subordonner définitivement

l'on sanctuarise- je reprends le mot car c'est le « vrai » mot-, le CHSCT, que l'on renforce ses moyens afin que ce lieu de sérénité- j'insiste sur ce terme -, dégagé des autres jeux internes de l'entreprise,

le prouve : une étude du cabinet APICIL Mozart Consulting indiquait récemment que le coût global du mal-être au travail se monte à 12 600 euros par an et par salarié du privé

par les entreprises si seulement elles prenaient en compte ce que cette étude appelle le désengagement salarié-employeur, qui peut se traduire par des arrêts causés par une charge de travail trop lourde, par des, par par des problèmes de santé et de sécurité ou du fait d'une perte de sens au travail, d'un manque de reconnaissance, d'information, de dialogue social, d'un isolement ou de conditions de

Une entreprise et des organismes peuvent décider de réunir régulièrement leurs instances ensemble. De ce point de vue, la proposition de Mme David me paraît frappée au coin du bon sens.

et ce parce que vous voulez qu'il y ait moins de représentants des syndicats et du personnel dans les entreprises, de la même manière que vous voulez moins d'élus locaux et moins de parlementaires. C'est une philosophie du pouvoir qui vise à renforcer en permanence l'exécutif, le décideur par rapport à ceux qui interviennent dans ce qu'on appelle les parties et qui doivent décider dans une entreprise comme dans la société.

produits chimiques, poussières fines, etc. Il y a d'énormes enjeux environnementaux. Il y a même d'énormes enjeux en termes de sécurité environnementale. Or le CHSCT est un lieu de vigilance collective en plus d'être celui de la prévention,

du travail de l'ensemble des représentants du personnel dans leurs différentes fonctions, et un objectif, qui me paraît aujourd'hui essentiel, de préservation d'un travail spécifique sur les problèmes de santé qui prennent de plus en plus d'importance et de gravité dans les entreprises. Vous avez entrouvert une porte, madame la ministre, en évoquant la possibilité de créer au sein du nouvel organe fusionné une sous-commission qui serait en charge des compétences actuelles du CHSCT. Pourquoi le Gouvernement ne prend-il pas l'engagement de rendre la constitution de cette cellule à l'intérieur du grand ensemble obligatoire et de droit ? Les objectifs

la ministre. Le coeur du sujet, c'est que nous croyons que lorsqu'il est à la fois social et économique, le dialogue apporte de la valeur. J'ai cité deux exemples, celui de la prévention des risques psychosociaux et, plus rapidement, celui des fusions-acquisitions. Je voudrais vous en donner deux autres.

Avec le comité social et économique, cette question sera traitée individuellement dans le respect du secret médical, mais l'aspect organisationnel, qui ne concerne jamais une seule personne,

des travaux de la commission des affaires sociales, le groupe socialiste a préféré, plutôt que d'évacuer l'ensemble de l'article 2,

scrutin est ouvert.

Quelle société voulons-nous ? N'en déplaise à l'ancien Premier ministre qui fustigeait « la société du farniente », le droit au temps libre est inscrit dans l'ADN du courant de pensée émancipateur auquel nous adhérons. Tout d'abord, je tiens à faire remarquer que, y compris à droite, l'idée des 32 heures rémunérées à équivalence temps plein a fait du chemin. Elle a même été appliquée : on peut penser à la loi Robien de 1996, qui, en l'échange d'exonération de cotisations sociales, permettait aux entreprises d'appliquer les 32 heures. C'est ainsi que des sociétés comme la Macif, Fleury Michon ou Télérama avaient sauté le pas.

En effet- on en vient au pur débat économique -, l'augmentation du temps libre est aussi une chance pour le développement de nouvelles activités économiques. pour appréhender concrètement l'intérêt des 32 heures hebdomadaires payées 35, il faut dresser un portrait précis de la société : la productivité par travailleur augmente en permanence, tout comme le chômage de masse. Par principe, la consommation et les besoins ne sont pas infinis, ce qui implique, à terme, la raréfaction de l'emploi. Un nouveau partage du temps de travail nous semble donc le meilleur moyen de lutter efficacement contre le chômage tout en maintenant le niveau de productivité par travailleur. C'est notamment le raisonnement qu'a suivi la Suède pour appliquer les 32 heures, après une première expérimentation par Toyota en 2002. Le résultat est clair : cette réforme a permis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

Les DUP concernent plus de 60 % des entreprises de 50 à 200 salariés disposant d'une instance représentative du personnel. D'après la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, 24 % des entreprises de 200 à 300 salariés ont une DUP. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un accord collectif majoritaire peut déjà procéder au regroupement des instances représentatives du personnel, qu'il s'agisse de deux d'entre elles ou des trois. L'instance ainsi créée exerce l'ensemble des attributions des institutions qu'elle regroupe en leur lieu et place. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, en application du code du travail issu de la loi du 17 août 2015, l'employeur peut mettre en place une DUP en y incluant le CHSCT. Mais il s'agit d'un en y incluant le CHSCT. Mais il s'agit d'un regroupement et en aucun cas d'une fusion. Au sein de la DUP, chaque institution- délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT -conserve ses attributions. Or la fusion ici proposée

d'alerte et d'analyse. Il doit conserver sa personnalité morale, la capacité à ester en justice. Enfin, il doit pouvoir recourir à des expertises spécifiques avec un financement dédié.

de négociation, l'accord collectif, l'accord d'entreprise, mais pour les instances représentatives du personnel, il n'y a pas le choix. L'obligation est faite à tous de se caler sur le même modèle et de fusionner l'ensemble

vous supprimez les commissions obligatoires incluses dans les comités d'entreprise. Comment pouvez-vous justifier, madame la ministre, la suppression de la commission de la formation professionnelle et de l'emploi alors même que la montée en charge des besoins en connaissances et en qualifications est importante, au vu des évolutions technologiques constantes ? Comment pouvez-vous également justifier la

mais de plus en plus difficile, au vu de la stagnation des salaires, de l'envolée des prix et de la pénurie de logements sociaux. Ainsi, vous proposez de supprimer des commissions nécessaires à à l'accès aux informations pour les salariés comme à la tranquillité des employeurs, lesquels, en jouant le jeu de la transparence, étaient insoupçonnables. Ces groupes de travail ont montré depuis leur création toute leur expertise et leur capacité à aiguiller les comités d'entreprise. L'amendement

Ces seuils, qu'il s'agisse de celui de onze ou de celui de cinquante salariés, constituent des freins psychologiques et administratifs au développement des entreprises et agissent comme des freins à leur croissance. Ils sont d'ailleurs dans les faits peu respectés. À titre d'exemple, seulement 38 % des entreprises de cinquante

Nous sommes bien évidemment opposés à un éventuel relèvement des seuils légaux, qui, d'ailleurs, ne semble pas faire partie de la concertation avec les organisations syndicales. Cette problématique recouvre les questions relatives non seulement aux attributions et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, mais également aux moyens, à la formation et au financement du recours aux expertises, qui, comme vous le savez, madame la ministre, est un sujet de fâcherie. Vous en avez l'illustration ici. C'est pourquoi

Il s'agit là du nombre de mandats successifs pouvant être accomplis par les délégués, à l'intérieur de l'entreprise.

l'on ne limite pas le nombre de mandats. En tout état de cause, on ne voit pas bien pourquoi nous devrions nous ingérer dans cette affaire, sauf à vouloir étendre aux délégués syndicaux ce qui a été décidé pour les élus de la Nation

de prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, si je peux m'exprimer ainsi : le cumul des mandats syndicaux. La commission a abondé dans son sens. les salariés ne s'engagent pas dans des mandats d'élus représentants du personnel ou dans des fonctions de délégué du personnel, c'est pour d'autres raisons que celles qui sont invoquées.

seraient affectés par ces discriminations. C'est en s'attaquant à ce problème que l'on renouvellera le vivier potentiel de délégués syndicaux et de représentants du personnel.

J'ai dit, par ailleurs, que nous allions prévoir des dispositions en matière de discriminations syndicales, qui, si elles sont rares, sont graves et, donc, non tolérables. En ce qui concerne les représentants du personnel élus, il s'agit d'éviter une surprofessionnalisation à vie.

le tout dans le cadre d'un choix relevant uniquement des élus. Un amendement présenté par notre rapporteur a permis une mise en concurrence des cabinets d'experts. Le présent amendement tend, en outre, à prévoir le partage de la charge financière des expertises entre l'entreprise et l'instance fusionnant les IRP, ainsi que la création d'un barème pour ces frais.

de l'article 2 du présent projet de loi, qui prévoit de réorganiser l'ensemble des institutions représentatives du personnel et de refondre également les règles de négociation. La fusion des CHSCT avec les autres instances représentatives du personnel inquiète tout particulièrement. Le CHSCT rempli en effet des missions très spécifiques. Il mène les enquêtes lors d'accidents du travail graves, il tient à jour le registre des accidents du travail et le document d'évaluation des risques, il donne des avis et interpelle l'employeur sur les risques dans l'entreprise, il peut faire suspendre en justice les réorganisations du travail et les restructurations qui portent atteinte à la santé physique et mentale des salariés, il peut inciter les salariés à exercer leur droit de retrait face à une situation de danger,

L'alinéa 3 porte un coup particulièrement grave à la compétence, aux pouvoirs des délégués syndicaux. Les dispositions concernées expriment la volonté du Gouvernement de permettre à l'instance unique de négocier directement des accords de groupe et ainsi de se substituer, dans cette fonction, aux délégués syndicaux. Le texte que vous proposez, madame la ministre, est, je l'ai déjà dit, imprécis. Il peut laisser présager un véritable coup de pouce contre les délégués et, par là même, contre les syndicats. M. Milon, président-rapporteur, souligne même, fort judicieusement, que l'étude d'impact n'aborde absolument pas ce point. Vous me direz que votre volonté est de pallier l'absence de délégués des nombreuses petites et moyennes entreprises. Ce que vous ne dites pas, en revanche, c'est que l'ensemble des entreprises, y compris les plus importantes,

entre le rôle de l'instance en tant que négociatrice des accords collectifs et celui des délégués syndicaux qui, dans ce cas de figure, seraient dépossédés d'une de leurs principales attributions. » Madame la ministre,

Les délégués syndicaux sont au coeur de la démocratie sociale, ils assurent la représentation syndicale. Leur remise en cause participe, de notre point de vue et nous ne sommes pas les seuls à porter cet état d'esprit, du véritable coup d'État social

lequel prévoit que l'instance unique peut exercer les compétences de négociation, et non qu'elles les exercent systématiquement par défaut, sauf accord majoritaire contraire. À travers À travers l'instance, on doit permettre d'envisager les mécanismes selon lesquels les compétences en matière de négociations collectives, en l'absence de représentants syndicaux ou lorsque les syndicats présents souhaiteront lui déléguer certaines missions, pourront fonctionner. Il s'agit de rendre le dialogue social plus efficace et de représenter de façon plus adéquate la collectivité de travail. Cette instance unique va le permettre. Le droit international rappelle le principe de la primauté des organisations syndicales pour négocier avec l'employeur ou les organisations d'employeurs.

dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l'employeur, notamment en vue de renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Or, nous le savons, l'instauration de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes n'est pas naturelle, mais passe par le développement de pratiques itératives, par le renforcement du service public éducatif pour élever le niveau global de qualification, par la construction de l'estime de soi et par l'émancipation. Ce projet s'inscrit dans le temps long et je suis convaincue que la participation de toutes nos concitoyennes à la vie collective de notre pays dans une association, une fondation, une coopérative et, bien sûr, dans l'entreprise, nous fera collectivement bénéficier de l'apport des parcours individuels. La discussion actuelle peut se résumer simplement : l'expérience des salariés peut-elle contribuer à moderniser le dialogue social et à améliorer la vie dans l'entreprise ? J'en suis convaincue, de même que de nombreux salariés et beaucoup de chefs d'entreprise. Le rétablissement de cet alinéa, complété par mes soins d'un deuxième engagement de société fondamental, à savoir le renforcement de l'emploi des personnes handicapées, est gage de réussite de la politique de l'entreprise dynamique et solidaire, de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de l'emploi des personnes en situation de handicap. Les salariés de genre féminin et les personnes qui vivent avec un handicap, quand il s'agit de femmes, souffrent toujours de fortes discriminations au travail, dans l'accès à l'emploi ou à des responsabilités, dans la reconnaissance de l'intérêt de leur travail au sein de l'entreprise, dans les relations de travail avec leurs collègues et avec leur hiérarchie. Ces sujets ne sont pas suffisamment portés dans le dialogue social courant dit « de droit commun ». Alors que la mixité de la réflexion est à même de réduire les biais qui freinent les avancées sociétales hautement profitables au dynamisme et à la modernisation de nos rapports humains dans tous les secteurs d'activité, particulièrement dans l'entreprise, où les idées reçues ont la vie dure, la participation des salariés aux discussions et à la prise de décision sur ces deux sujets ne réglera pas l'ensemble des problèmes, mais constitue un élément nécessaire pour lutter contre les discriminations insidieuses et souvent involontaires

Il s'agit, vous l'aurez constaté, d'un amendement de repli. J'ai bon espoir que notre assemblée, dans sa sagesse, adhère à l'esprit de mes propositions ! Si l'argument de promotion pour les représentants du personnel du renforcement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne retenait pas votre adhésion, cet amendement de repli tend à conférer la possibilité de déterminer les conditions dans lesquelles les représentants du personnel seront mieux associés aux décisions de l'entreprise en vue de renforcer l'emploi des personnes handicapées. Il vise donc à donner de l'élan pour satisfaire, de façon harmonieuse et consentie, aux obligations issues de la loi de 2005, à savoir 6 % de salariés avec handicap dans les effectifs d'une entreprise, fut-elle privée ou publique. Souvent, les frilosités, les idées reçues, des pudeurs inappropriées ou des préjugés freinent le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

qui, ayant des besoins spécifiques, n'en ont pas moins des compétences professionnelles et des capacités relationnelles et organisationnelles utiles à l'entreprise. Le dialogue social doit prendre en charge cette question de progrès social, qui, par ailleurs, fait l'objet d'une priorité du Président de la République, lequel a souhaité que soit développée une politique inclusive des personnes handicapées. Cette politique inclusive doit véritablement irriguer l'ensemble des politiques publiques, et particulièrement la politique de l'emploi.

a supprimé cet alinéa au nom du principe de non-discrimination. Pourtant, alors même que l'article 2 a pour objet d'améliorer les conditions du dialogue social dans les instances représentatives du personnel,

des sujets qui intéressent directement la gestion de l'entreprise : organisation du travail, formation professionnelle, gestion économique et financière, etc. En effet, nos entreprises restent majoritairement organisées sur un modèle de division des tâches et de séparation entre la prise de décision par les dirigeants et son application par les salariés. Or, l'entreprise étant également un bien collectif, il apparaît nécessaire d'en moderniser la gouvernance. Si toutes les questions sociales qui concernent les salariés sont remises à plat dans ce projet de loi et, demain, dans les ordonnances qui en seront issues, il n'y a aucune raison d'exclure du nouveau cadre de relations entre salariés et employeurs les choix économiques qui ont trait à la vie de l'entreprise. Mieux encore, ce partage de la prise de décision permettrait de sauver certaines entreprises de décisions regrettables. Nous connaissons tous des exemples de choix économiques désastreux et douteux, faits unilatéralement par des directions d'entreprise sous pression des actionnaires. Si les salariés pouvaient intervenir réellement dans les décisions économiques de l'entreprise ou du groupe, il est certain que beaucoup d'emplois seraient sauvés. Dans le Pas-de-Calais, par exemple, deux sites de l'industrie

internationaux de l'industrie papetière, désireux de diminuer la production en Europe pour faire remonter les cours du marché et délocaliser les productions hors d'Europe. Notre amendement vise donc à mieux associer les représentants de salariés

aux décisions de l'employeur dans certaines matières, notamment pour renforcer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il s'agissait de renforcer la présence salariale et, donc, la transparence et la confiance, en permettant aux salariés ou à leurs représentants de participer à la gouvernance. Cet alinéa a été supprimé par la commission des affaires sociales, au motif que son imprécision pourrait porter atteinte à la liberté d'entreprendre et pourrait se traduire par des mesures préjudiciables à la capacité de l'employeur à diriger son entreprise. Parce qu'il nous semble nécessaire de mieux prendre en compte le point de vue du personnel dans les processus de décision stratégique de l'entreprise, nous proposons tout simplement de rétablir cet alinéa.

aux auteurs de ces amendements. Je me réjouis que la promotion du dialogue social, la réforme des IRP et leur simplification, introduisant plus de lisibilité et d'efficacité pour les employeurs et les salariés, soient ainsi débattues avec sérénité dans notre assemblée. dans notre assemblée. Notre commission des affaires sociales a apporté son soutien à la création d'une instance unique fusionnant les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Elle a fait preuve d'une volonté réformatrice plus marquée que celle du Gouvernement, en prévoyant que cette nouvelle instance serait dotée de droit d'une compétence en matière de négociation des accords d'entreprise. Elle a également supprimé des habilitations demandées par le Gouvernement. Elles étaient, selon nous, trop imprécises- c'est le cas de celle qui prévoyait une meilleure association des représentants des salariés aux décisions de l'employeur -ou semblaient entretenir une instabilité juridique néfaste à la bonne gouvernance des entreprises, s'agissant de la représentation des salariés dans leurs conseils d'administration, dont la dernière réforme, par la loi Rebsamen en 2015, n'est pas encore complètement applicable.

La commission sollicite le retrait de l'amendement n° 207 rectifié de Mme Lamure, dès lors que le Gouvernement aura pu nous préciser ses intentions sur les questions de seuils.

aux représentants du personnel en matière de recrutement, ce qui pourrait être contraire au principe de non-discrimination, alors que ces deux thèmes font déjà l'objet d'une négociation annuelle obligatoire. Le groupe CRC, au travers de ses amendements n 107 et 108, propose même de mettre en place une véritable cogestion des entreprises. Ce serait aller, selon la commission, à l'encontre de la liberté d'entreprendre et du pouvoir de direction de l'employeur.

et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou CHSCT. Dénoncée par nombre de nos collègues, que je rejoins sur cette fusion entraînera inévitablement un affaiblissement des prérogatives des représentants du personnel dans les entreprises et une réduction des moyens qui leur sont dédiés. Écologiste de coeur et de conviction, je tiens à souligner le véritable danger que représentent ces mesures pour la santé et la sécurité des travailleurs. La fusion des instances représentatives du personnel va reléguer ces thématiques, pourtant ô combien importantes, au second plan. au sein de la future instance unique, les prérogatives des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vont certainement se retrouver submergées par une multitude d'autres sujets. Si l'on défend un droit du travail véritablement moderne et respectueux des salariés, c'est au contraire un renforcement, et même un élargissement, des compétences du CHSCT qu'il faudrait prévoir dans la loi

des CHSCT à la prévention en santé globale, pour le bien-être au travail et dans la vie quotidienne, mais aussi à la protection de l'environnement

la violence de la révolution du travail, sa rapidité laissent dans des zones grises une multitude de maladies qui ne sont même pas encore complètement répertoriées ni identifiées comme étant dues au travail et aux nouveautés au sein

Assumez ce choix-là ! Il est mauvais, on vous le dit. Mais assumez-le ! Ne nous faites pas croire le contraire avec des envolées langagières, cela ne tient pas la route

Watrin, pour explication de vote.

pas cogérée. Cette codétermination donne en tout cas un vrai pouvoir aux organisations syndicales. Par ailleurs, pour des raisons historiques- je ne suis pas sûre qu'il faille toujours comparer -, le syndicalisme allemand n'est pas pluraliste. Il n'existe souvent qu'un seul syndicat

La commission a souhaité que cette compétence de négociation soit exercée de plein droit par l'instance ; libres aux partenaires sociaux dans l'entreprise de refuser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

les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d'administration et de surveillance des sociétés dans le cadre des seuils mentionnés aux articles L. 225-27 et L. 225-79-2 du code de commerce,

Avec cet amendement, le Gouvernement précise qu'il ne souhaite pas modifier le champ des entreprises concernées. Dont acte. Nous aurions préféré que cette incertitude soit levée plus tôt. Le Gouvernement souhaite également renforcer la formation des représentants des salariés siégeant dans ces conseils. Nul ne peut s'y opposer. Il y a d'ailleurs plus simple qu'une ordonnance pour le faire : j'invite Mme la ministre à prendre un décret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

Mis en place sur une plus grande échelle, ce dispositif pourrait toutefois contribuer à rapprocher davantage les salariés de leurs syndicats et les inciter à s'engager dans le dialogue social d'entreprise. Toutefois, l'absence d'évaluation ou de précisions sur ce point dans l'étude d'impact oblige à s'en tenir

vote. Madame la ministre, je suis bien évidemment favorable à l'amendement du Gouvernement visant à renforcer et à simplifier l'accès à la formation économique, sociale et syndicale des représentants des salariés. Je souhaite profiter de ce débat pour encourager le Gouvernement à se pencher à cette occasion d'autres ministères, sur la formation au dialogue social des cadres et des managers d'entreprise. Même si des progrès sont observés ici ou là dans les universités ou les grandes écoles, peu de place est accordée au dialogue social dans les cursus de formation consacrés au management. Les partenaires sociaux avaient déjà souligné cette carence lorsque, en 2011, j'avais rédigé avec notre ancien collègue Joël Bourdin un rapport d'information sur la prospective sur le pacte social dans l'entreprise. Plus récemment, en mai 2016, un avis du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, soulignait que ni la formation initiale ni la formation continue ne sont encore à la hauteur des besoins. Le CESE relève en effet que, même dans les enseignements où l'on peut s'attendre à trouver une formation au dialogue social, comme les masters spécialisés en ressources humaines, le dialogue social paraît souvent se limiter à un module de formation juridique sans prendre en compte les retours d'expérience ou les études de cas, et laisse peu de place à l'intervention des partenaires sociaux dans ces formations. Madame la ministre, puisque nous sommes réunis autour du « renforcement du dialogue social », je vous engage à explorer avec votre collègue ministre de l'enseignement supérieur toutes les pistes de nature à former au dialogue social les futurs responsables et dirigeants, avec la participation et l'intervention des partenaires sociaux dans ces formations. J'irai même plus loin pour que la culture du dialogue social « infuse » toute notre société, il faudrait que nos jeunes y soient sensibilisés durant toute leur scolarité, chaque fois qu'une occasion se présente. Je pense en particulier au stage de troisième, aux fonctions de délégué de classe ou, au-delà

À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement appelant le Gouvernement à le redéfinir plutôt qu'à le renforcer. La commission des affaires sociales a supprimé

lorsque le propriétaire de plus de 50 % des parts sociales d'une entreprise décide de les vendre. Ce droit de préemption concernerait les entreprises de moins de 250 salariés. Cette proposition se situe dans le prolongement de la loi dite Hamon de juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui créait un droit d'information des salariés au moment de la cession de l'entreprise. l'entreprise. C'est une proposition d'intérêt général pour lutter contre le chômage. Il s'agit de privilégier la reprise de l'entreprise par ceux qui ont à coeur la préservation de l'emploi, de tous les emplois, au contraire des repreneurs qui considèrent systématiquement l'emploi comme une variable d'ajustement pour assurer un taux de profit acceptable pour les actionnaires. M. Retailleau parlait tout à l'heure de lutter contre le chômage : nous vous invitons, mes chers collègues, à voter cet amendement qui tend à créer les conditions pour permettre une décision réfléchie et responsable des salariés. En effet, lorsqu'un employeur trouve un acquéreur, il doit le notifier aux salariés, les informer du prix et des conditions de la vente et leur donner un accès aux documents comptables. Pendant deux mois, les salariés pourront se substituer au nouvel acquéreur et devenir propriétaires propriétaires de l'entreprise. Je l'ai souligné, c'est une proposition d'intérêt général, qui vise à replacer l'emploi au coeur des préoccupations économiques en s'appuyant sur de nouveaux droits pour les salariés. La modernité, le progrès, c'est cela, et non la soumission accrue des travailleurs à l'actionnariat que porte votre projet

l'économie sociale et solidaire. Je ferai deux remarques. Premièrement, aucune disposition dans le texte n'aborde cette question, et pour cause : il s'agit d'une disposition relevant du code de commerce et non du code du travail. Deuxièmement, le droit de préemption au profit des salariés

Enfin, je rappelle que la procédure de recherche d'un repreneur prévoit déjà à l'article L. 1233-57-10 du code du travail une information spécifique de l'employeur à destination des salariés qui souhaitent déposer une offre de reprise sous la forme notamment d'une société

dans les conseils d'administration des entreprises est un atout en matière sociale, mais aussi stratégique. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui une série de mesures législatives qui doivent permettre à notre modèle de continuer sa réorientation en abaissant à 500 le seuil à partir duquel la présence d'administrateurs salariés est requise, seuil valant tant dans les sociétés et leurs filiales dont le siège social est fixé sur le territoire national que dans celles dont le siège social est à l'étranger. Il apparaît judicieux de permettre à un projet de loi d'habilitation destiné à renforcer le dialogue social de développer une forme de représentation et de participation des salariés qui favorise le dialogue social, et donc la performance des entreprises. La parole est à M. David Assouline, pour présenter

De fait, la présence des salariés dans les conseils d'administration des entreprises constitue, en toute hypothèse, un atout en matière sociale, mais aussi en termes de stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin dans l'extension de la présence des administrateurs salariés pour accroître la diversité des profils au sein des conseils d'administration, non plus pour instituer un modèle qui consacre la suprématie de l'actionnaire dans la gestion de l'entreprise, mais bien pour instaurer un cadre au sein duquel la gouvernance d'entreprise favorise l'investissement de long terme. En conséquence, le premier amendement qui vous est proposé vise à abaisser à 500, pour les entreprises dont le siège social est en France, le seuil déclenchant la présence de deux administrateurs salariés et à 5 000 ce même seuil pour les entreprises dont le siège se situe à l'étranger. Ces amendements

Le seuil d'effectif initial- 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France -a été abaissé à peine deux ans plus tard par la loi Rebsamen du 17 août 2015- 5 000 salariés en France et à l'étranger ou 1 000 en France -, qui a également supprimé une dérogation qui bénéficiait aux holdings. La loi Rebsamen avait prévu une période transitoire pour la mise en application de ce nouveau seuil : les entreprises nouvellement soumises à cette obligation ont jusqu'à courant de l'année 2018 pour se mettre en conformité avec elle. Il semble donc bien prématuré de généraliser ce régime à toutes les entreprises comptant au moins 500 salariés. Outre Outre que l'équilibre de la gouvernance d'entreprises de taille moyenne serait bouleversé, cette disposition aggraverait l'instabilité juridique autour de la représentation des salariés dans les conseils d'administration qui est entretenue depuis 2013. Or de quoi ont actuellement besoin nos entreprises si ce n'est d'un cadre juridique stable pour se concentrer sur le développement de leur activité ? La commission des affaires sociales a supprimé l'habilitation que le Gouvernement souhaitait obtenir dans ce domaine, notamment parce que celui-ci n'a jamais précisé, au moins jusqu'à ce soir,

Nous proposons qu'il y ait au moins deux administrateurs salariés dans les entreprises de 500 à 1 000 salariés ; dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, ce nombre serait au moins égal au tiers, sans pouvoir être inférieur à Cette proposition, qui va dans le sens de celle qui a été défendue par les syndicats, permettrait, avec l'amendement présenté plus en amont, d'harmoniser nos pratiques avec celles de nombreux pays européens.

Ces amendements tendent à modifier cette logique en fixant le nombre de représentants des salariés en fonction de la taille des entreprises, le portant au tiers des conseils dans les plus grandes entreprises. Il est articulé avec l'amendement n° 154 rectifié , qui vise à abaisser le seuil d'effectifs à partir duquel la représentation des salariés est obligatoire dans les conseils d'administration et que nous avons rejeté.

exprimer une opinion différente de celles qui viennent d'être exposées au sujet de la mutation de la gouvernance d'entreprise.

Ce qui pose problème avec ces amendements, que nous allons repousser, c'est qu'ils tendent à créer dans la loi une obligation à la place d'un dialogue social.

La représentation des salariés au sein des conseils d'administration est très insuffisante en France, car elle est limitée aux seules très grandes entreprises.

En clair, le plafond actuellement applicable deviendrait un seuil plancher. À l'évidence, une telle disposition constituerait un saut qualitatif indéniable

: « [ ...] le poids des actionnaires doit être équilibré, en privilégiant ceux qui jouent le long terme et en donnant la parole aux autres parties prenantes de l'entreprise. » C'est ce que vient de rappeler notre collègue Jean Desessard.

Si cet article prend déjà en compte les cas de discrimination à l'embauche ou à l'exercice d'activités, il ne fait que couvrir une part limitée des cas de discrimination dans le monde du travail. En effet, comme l'ont relevé successivement

Si la justice a déjà rendu des jugements contre des entreprises responsables de discrimination, les juges n'ont à l'heure actuelle aucune base légale solide sur laquelle s'appuyer. Ainsi le jugement ne tient-il que sur l'interprétation de l'article 225-2 du code pénal. On pense ici, par exemple, au groupe La Poste, à la SNCF ou à l'entreprise Ikea, condamnés ces dernières années pour avoir dévalué des salariés au motif qu'ils avaient des responsabilités syndicales. Malheureusement, en l'absence de base légale solide, ces jugements peuvent être facilement cassés à l'occasion d'un second recours. Par ailleurs, à la difficulté de définition par le juge de ce qu'est une discrimination syndicale s'ajoute la question du taux de non-recours, favorisé justement par ce sentiment que la loi n'est pas appliquée. Comme le disait à juste titre Simone Veil, « lorsque l'écart entre les infractions commises et celles qui sont poursuivies est tel qu'il n'y a plus à proprement parler de répression, c'est le respect des citoyens pour la loi, et donc l'autorité de l'État, qui sont mis en cause ». Au final, cet amendement vise à mettre en application les recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, qui déplorait en juin 2016 les actes de représailles contre les représentants syndicaux signalés » et engageait la France à prendre des mesures efficaces en matière de protection des personnes engagées dans des activités syndicales, de prévention et de répression de toutes les formes de représailles. Ainsi, les dix-huit experts de l'ONU ont considéré que la France sous-estimait la répression syndicale, alors même que la jurisprudence a tenté, de manière incomplète, de donner un cadre juridique à la répression des actes de discrimination. À ce titre, on ne peut que saluer l'arrêt de la Cour de cassation de janvier 2015, aux termes duquel le cas d'un salarié du secteur privé disposant de mandats syndicaux qui ne bénéficie d'aucun entretien d'évaluation depuis plusieurs années et ne connaît aucune évolution de carrière laisse

Cet amendement s'inscrit donc dans cette dynamique en visant à sécuriser le parcours des salariés engagés, alors même que la crainte de représailles est le premier motif de non-engagement syndical.

je ne comprends pas très bien à quoi correspond le « refus d'une classification », la troisième modification proposée dans l'amendement -est déjà sanctionné s'il a pour motif les activités syndicales du salarié concerné, qui peut donc se tourner vers le juge.

tout motif basé sur cette même action. L'amendement vise également à protéger l'ensemble des salariés qui seraient susceptibles de produire des preuves ou témoignages lors de la procédure judiciaire. Il tend ainsi à apporter une protection permettant l'accès libre à la justice, libérant les parties demanderesses de toute entrave professionnelle uniquement motivée par la mise en oeuvre de ladite procédure. Au fond, il s'agit simplement de donner force de loi à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, rappelée encore en février dernier, aux termes de laquelle le droit d'ester en justice est une liberté fondamentale conférée à tout salarié, qui doit pouvoir s'exercer sans restriction. Ainsi, les juges ont toujours annulé les licenciements pris sur ce motif. De la même manière, ils ont, par exemple, considéré que doit être annulé un licenciement motivé par le témoignage en justice d'un salarié en faveur d'un ancien collègue. Dans le même sens, il a été jugé que, sauf mauvaise foi de la part du salarié, le dépôt d'une plainte constituait l'exercice d'un droit et ne pouvait pas être une faute justifiant un licenciement. La loi devant être une protection supplémentaire, nous vous proposons d'inscrire très clairement ces dispositions dans le code du travail.

le 14 octobre 2015, relative à la protection des salariés ayant intenté une action en justice à l'encontre de tout membre de leur entreprise, société ou groupe, mais qui n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour ; on peut le regretter, mais c'est ainsi.

ou licenciement. Un salarié ou candidat à l'embauche victime d'une sanction pour avoir subi ou dénoncé des faits de discrimination, ou de harcèlement social ou moral, est protégé de la même manière. En outre, dans les cas qui ne relèveraient ni de la discrimination ni du harcèlement, le juge peut remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement. Une sanction infligée à un salarié pour des motifs similaires encourrait l'annulation par le juge pour absence de motif valable de la sanction.

libellé : La parole est à M. Christian Favier. L'exercice du mandat syndical se heurte souvent, on le sait, au manque de temps des salariés pour s'informer sur leurs propres droits. Pourtant, le premier rôle des représentants des salariés est de rester en contact avec leurs collègues pour faire remonter les problèmes dans les instances correspondantes, mais aussi pour les informer des décisions prises, de leur impact et de leurs conséquences sur les conditions de travail de chacun. Les administrations publiques, quant à elles, ont le dispositif de l'heure de délégation syndicale, qui permet aux syndicats et aux salariés de prendre une heure pour échanger sur les points qu'ils souhaitent. Cette respiration est indispensable pour la vie syndicale dans nos établissements scolaires, nos collectivités, nos hôpitaux, pour que les agents puissent vraiment avoir accès aux informations les concernant. Ne serait-elle pas utile, aussi, dans le secteur privé ? Madame la ministre, la mise en oeuvre de la délégation unique du personnel, la DUP, se soldera par une baisse du nombre d'élus et du nombre d'heures de délégation, et par une raréfaction des réunions. Quelle crédibilité accorder au débat que nous venons d'avoir sur l'article 2 si nous ne créons pas les conditions pour que l'expression des salariés puisse avoir lieu dans l'entreprise ? À l'Assemblée nationale, le rapporteur a argué que les salariés avaient toujours le droit de se réunir en dehors du temps de travail et que les délégués pouvaient aller et venir dans l'entreprise pour discuter. Plus grave encore, cette heure mensuelle pourrait, selon lui, désorganiser le travail de toute l'entreprise. Mes chers collègues, il est temps d'améliorer partout l'information des salariés en instaurant, comme nous le proposons, cette heure d'information syndicale dans toutes les entreprises.

Il prévoit, tout d'abord, de créer une heure mensuelle d'information syndicale à laquelle les salariés seraient autorisés d'assister sur leur temps de travail, sur le modèle de dispositions similaires qui existent dans la fonction publique. à procéder à deux autres modifications visant à élargir le droit d'information des salariés : il leur donne accès à la base de données économiques et sociales, la BDES, de l'entreprise lorsqu'une offre de vente leur est faite et ouvre, dans ce cas, une nouvelle possibilité de faire appel à un expert-comptable aux frais de l'employeur. Il me semble que, dans ce cas précis, notre assemblée peut se rallier à la sagesse de nos collègues députés. La BDES doit être réservée à l'information des instances représentatives du personnel en vue de la préparation de leurs avis, tandis qu'il n'est pas souhaitable d'imposer dans chaque entreprise cette heure d'information syndicale, qu'elle est libre,

parfois que des entreprises n'embauchent pas pour l'unique raison qu'elles ne souhaitent pas franchir un seuil qui impliquerait de nombreuses contraintes administratives et un surcoût de certaines cotisations sociales. Nous connaissons tous des entreprises qui ne veulent pas passer de 49 à 50 salariés. Bien sûr,

Bien que l'on puisse partager pleinement la philosophie de cet amendement, nous ne pouvons que constater qu'il est contraire à la Constitution. Plus spécifiquement, il est contraire à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel relative à la recevabilité des initiatives parlementaires en matière de recours aux ordonnances. Par deux décisions, l'une du 20 janvier 2005 et l'autre du 31 juillet 2014, il a interdit

Merci, mon cher collègue et le projet de loi organique pour la régulation de la vie publique, d'autre part, il va être procédé à la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires. Les listes des candidats ont été publiées ; je n'ai reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu